La séance est reprise. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande d'avancer l'examen des quatre conventions internationales en procédure simplifiée et du projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée, initialement prévu jeudi 27 octobre matin, au mercredi 26 octobre après-midi à l'issue de l'examen du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Si nous terminons l'examen de ce texte dès ce soir, ce qui semble possible, les conventions internationales seront examinées à l'issue des questions d'actualité au Gouvernement. Par conséquent, nous ne siégerions pas jeudi. Acte est donné de cette demande. En conséquence, nous pourrions avancer le délai limite d'inscription des orateurs dans la discussion générale du projet de loi autorisant Il n'y a pas d'opposition ? ... Il en est ainsi décidé. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 53 au sein de l'article 2. Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

votre credo, et tant pis pour la précarisation croissante ! Par cet amendement, nous proposons au contraire de renforcer les malus pour qu'ils aient un effet réellement dissuasif, en augmentant les cotisations versées par l'employeur au régime d'assurance chômage et en les modulant en fonction de la durée des contrats. Il nous paraît justifié d'imposer une majoration des cotisations sociales des entreprises qui ne respectent pas le code du travail en abusant des contrats courts.

d'accélérer la transition écologique et sociale des grandes entreprises, nous proposons dans cet amendement, uniquement pour les multinationales, un mécanisme de malus calculé en fonction des objectifs de transition écologique, d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de relocalisation et de maintien de l'emploi.

comportement. Le Gouvernement a reculé chaque fois qu'un dispositif a été mis en place et a même allégé la fiscalité des entreprises. Ainsi, d'un côté, le Gouvernement a instauré le mécanisme de bonus-malus et, de l'autre, il a allégé la fiscalité des contrats courts. Jusqu'en avril 2019, le taux de la cotisation patronale d'assurance chômage était majoré de 0,5 point pour les CDD d'usage de quelques heures ou jours dans certains secteurs.

n° 89 rectifié. Pour faire passer la baisse inédite des droits des travailleurs privés d'emploi, le Gouvernement a prétendu équilibrer la réforme en instaurant un bonus-malus à destination des entreprises recourant abusivement aux emplois très courts,

Or les secteurs retenus dans le cadre du bonus-malus sont précisément visés, parce qu'ils se caractérisent par un taux de séparation au moins une fois et demie supérieur à celui des autres secteurs. En conséquence, le bonus conduit à des baisses du taux de cotisation patronale quand bien même l'entreprise reste à des taux de séparation anormaux par rapport à ceux des entreprises de secteurs bien plus vertueux., ce système illogique conduit à récompenser les « moins mauvais élèves » des sept secteurs engendrant 37 % des séparations.

Par cet amendement, nous proposons d'autoriser les Urssaf à ne communiquer aux entreprises que les données nécessaires au calcul du bonus-malus et non les données personnelles. Cela permettrait de concilier l'objectif de transparence vis-à-vis des entreprises dans la fixation de leur taux de contribution à l'assurance chômage, d'une part, et le respect de la vie privée de leurs anciens salariés,

le plein emploi -, le temps partiel et le halo du chômage. Selon l'Insee, en 2020, un peu plus d'un million de femmes étaient concernées par le halo du chômage, contre 866 000 hommes. En outre, les femmes sont deux fois plus touchées par le sous-emploi que les hommes. En 2019, 7,8 % des femmes actives étaient sous-employées contre 3,1 % des hommes. Enfin, en 2019, 28,4 % des femmes actives travaillaient à temps partiel. De plus, lorsqu'elles travaillent, les femmes perçoivent en moyenne une rémunération inférieure de 28,5 % à celle des hommes.

Ce serait une manière plus vertueuse d'utiliser une mesure incitative que de simplement conditionner l'octroi du bonus- comme c'est actuellement le cas -à un moindre recours aux contrats courts dans des secteurs déjà sinistrés par des taux de remplacement élevés.

par la volonté de réduire le taux de séparation. La réintégration de ce dispositif relance donc une expérimentation qui n'a fait l'objet d'aucune évaluation,

pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. En effet, même si le contrat est d'une durée plus longue, il maintient le travailleur dans une situation de précarité, ce qui va à l'encontre de la volonté affichée du Gouvernement lors de la mise en place du bonus-malus. Le maintien d'un CDD, même long, est source de désavantages pour le salarié, notamment pour conclure un bail ou un emprunt, et peut être source de stress et de souffrance au travail pour le salarié bloqué dans une précarité permanente. Aussi, par cet amendement, nous proposons de supprimer cet article afin de ne pas relancer un dispositif qui n'a fait l'objet d'aucune évaluation. Quel est l'avis de la commission ? Cet article,

Cette mesure, présentée comme devant limiter le recours aux contrats courts, légitime en réalité une forme de contrat aux droits réduits qui pourrait concurrencer le CDI et devenir une nouvelle norme. Privés d'indemnités de précarité, les intérimaires en CDII voient souvent leurs conditions de travail se dégrader. La preuve en est

: La parole est à Mme Céline Brulin. Cet amendement vise à encadrer le recours au travail temporaire en limitant le nombre de personnes employées en contrat d'intérim à 10 % de l'effectif total des entreprises comptant au moins onze salariés.

augmente de façon très significative d'année en année, tout particulièrement ces dernières années ; cela veut bien dire qu'il existe des besoins structurels de recrutement dans les entreprises.

Pourquoi une telle modification ? Pour les salariés de l'usine Proma de Gien, dans le Loiret, qui ont été injustement privés de leur prime supralégale et, à

dans le cadre d'un plan de restructuration, il était convenu qu'une indemnité de licenciement supralégale d'un montant de 23 000 à 35 000 euros serait versée aux salariés licenciés. Un an plus tard, la société se trouvait en cessation de paiements et placée en redressement judiciaire.

n° 96 du Gouvernement, monsieur le ministre,

qui nous sont le plus chers représente l'essence même du don : le don de son temps, le don de son énergie, le don de son quotidien. Mais se donner ainsi à l'autre ne doit pas signifier perdre perdre ses projets, ni perdre son temps, ni perdre sa trajectoire professionnelle. C'est tout l'objet de la validation des acquis de l'expérience : assurer à nos concitoyens que toute expérience de vie peut être pour eux une source de compétences, que ces compétences seront valorisées et constitueront une chance pour l'avenir.

« bloc de compétences » d'une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles. Pour rappel, un « bloc de compétences », notion introduite par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, son avenir professionnel, est défini comme un ensemble homogène et cohérent de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées évaluées et validées. Sur le papier, c'est beau, monsieur le ministre ; vous avez abondé dans ce sens devant l'Assemblée nationale, en vantant les mérites de la VAE : cette démarche serait moins longue, moins coûteuse, plus accessible et susceptible de redonner à une personne

que « la construction des blocs pourrait, sans une régulation d'ensemble, conduire à une amplification du flou des compétences et des savoirs des individus sur le marché du travail, avec un risque fort

des expériences hors de l'Union européenne. En principe, l'unique critère pour obtenir une VAE est d'avoir exercé pendant au moins un an une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec le contenu de la certification envisagée,

sans distinction, sont concernés par l'ouverture de la validation des acquis de l'expérience. L'accompagnement personnalisé et le financement des parcours de VAE sont accessibles aux Français de l'étranger, qui peuvent donc s'y engager. Le risque,

En première lecture, l'Assemblée nationale a profondément modifié l'organisation de la VAE, la transférant du code de l'éducation vers le code du travail dans un prétendu souci de simplification, renvoyant au règlement le soin de préciser les modalités d'organisation et de composition des jurys de validation des acquis de l'expérience. Cette modification censée introduire plus de souplesse et réduire les délais de certification risque pourtant d'éloigner ces jurys du monde universitaire, qui sanctionnait jusqu'alors la délivrance des diplômes en validant une expérience professionnelle équivalente. Le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a vu ses effectifs et ses moyens s'étioler au fil des dernières années, ne saurait être tenu pour responsable des retards pris dans l'organisation des jurys de VAE et se voir dépossédé de la mission de délivrance Il convient de s'assurer que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche resteront majoritaires dans la composition de ces jurys et que les règles de nomination demeureront

pour préparer la VAE et participer à la session d'évaluation devant le jury. L'Assemblée nationale a décidé d'allonger cette période de congé à quarante-huit heures. Je vous propose de le porter à soixante-douze heures pour permettre aux candidats de passer leur examen dans des conditions optimales.

Son principe est de rendre concomitants les processus d'acquisition des compétences par l'emploi et la formation, d'une part, et de reconnaissance des compétences, de l'autre. Alors que la VAE de droit commun suppose que l'expérience soit acquise antérieurement au démarrage de la procédure, nous souhaitons expérimenter une VAE permettant à des personnes de s'engager dans un parcours de montée en compétence progressif, alliant emploi et formation. Ce parcours serait accompagné, du début jusqu'à la fin, afin que le bénéficiaire rédige un dossier de validation des compétences acquises, c'est-à-dire progressivement au cours de ses périodes d'emploi et de formation. Les compétences seront alors sanctionnées par un jury de VAE. L'objectif est de tester des parcours sans couture et individualisés entre emploi et formation, qui supposent l'engagement de l'employeur aux côtés du salarié, afin de l'accompagner vers la certification et l'emploi durable. Ciblant les secteurs en tension, la VAE inversée est une nouvelle forme d'acquisition des compétences mieux adaptée aux besoins des entreprises et des secteurs d'activité, mais également aux personnes ne personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas s'engager dans un parcours de formation classique. La méthode est d'expérimenter pour tester la pertinence de ces parcours nouveaux dans les secteurs en tension. Afin d'asseoir juridiquement cette approche, le contrat de professionnalisation apparaît le plus adapté, car il allie périodes en entreprise et périodes en formation. Il offre également l'avantage de la sécurité, pour le bénéficiaire comme pour son employeur, et permet le financement des frais pédagogiques comme la perception d'un salaire.

n° 38 rectifié. Nous proposons la suppression de cet article pour contester le principe même de la gouvernance par ordonnances. Le recours systématique aux ordonnances par le Gouvernement démontre sa volonté de légiférer sans le Parlement. C'est un déni complet de ce qu'est le Parlement, c'est-à-dire un lieu de débats et d'échanges et non une simple chambre d'enregistrement.

de loi. La suppression de quinze ordonnances au sein de cette liste, effectuée par la commission des affaires sociales, aurait pour effet de rendre caducs des textes qui ont régi la situation de millions de personnes au cours de la période récente. Cette caducité entraînerait la disparition rétroactive de la base légale des modifications ayant été été introduites pour gérer ces situations, notamment pendant la crise sanitaire. Cela fragiliserait ces situations, qu'il s'agisse de celles de salariés, de demandeurs d'emploi ou d'entreprises. Le Gouvernement entend donc rétablir une liste quasi identique à la liste initialement prévue, la seule différence étant la suppression de la référence à l'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19, devenue sans objet à la suite de la décision du Conseil d'État du 19 mai 2021. Quel est l'avis de la commission ? Dans la logique

Lubin. Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement concernant les effets de la réforme de l'assurance chômage sur les jeunes. La réforme présentée par le Gouvernement va, une fois encore, produire un effet négatif pour deux catégories de personnes

Pôle emploi va prendre en compte sa période d'inactivité de six mois à cause d'un job ponctuel, ce qui va faire mécaniquement baisser le montant de son allocation. Alors que la vie chère, l'inflation et le chômage pèsent lourdement sur les jeunes, la réforme proposée par le Gouvernement risque de précariser un peu plus encore des personnes en situation difficile. C'est pourquoi

Mme Raymonde Poncet Monge. Dans une étude, l'économiste Yann Algan démontre que la réduction des indemnités de chômage présente des externalités négatives en matière de maintien de la masse salariale. Selon lui, « il existe aujourd'hui des arguments solides à la mise en place d'indemnisations chômage généreuses. chômage permet aux chômeurs de rejeter les propositions d'emploi de piètre qualité. Réduire la générosité de l'indemnisation pourrait donc se traduire par une diminution de la masse salariale. Ces conclusions se combinent à des centaines d'autres études évaluées dans la méta-analyse de la Dares, qui concluent que la baisse des taux de remplacement, la hausse de la durée d'affiliation et la diminution du temps d'indemnisation poussent les demandeurs d'emploi à accepter des emplois ne répondant pas à leurs aspirations. Un double phénomène se dessine : pour les chômeurs, la baisse des indemnités réduit leur capacité d'arbitrage afin d'obtenir des emplois de qualité et correctement rémunérés ; en retour, cela impacte la capacité des salariés en poste à négocier de meilleures conditions de travail et de rémunération, d'autant que des réformes antérieures ont déjà fragilisé leur propre faculté de négocier. Il est donc plus que probable que cette mécanique entraîne pour l'ensemble des salariés des métiers dits « en tension » une pression à la baisse sur les salaires et les avancées de carrière. Il est nécessaire d'obtenir des données solides sur les potentielles externalités négatives de la première réforme. Un rapport doit éclairer le Parlement sur les effets de la réforme de l'assurance chômage de 2019 sur l'évolution des salaires en France. Quel est l'avis de la commission ? Même argumentation que

». l'article 1, le Gouvernement souhaite en effet que le Parlement lui signe un chèque en blanc jusqu'au 31 décembre 2023 pour réformer l'assurance chômage après une simple consultation des partenaires sociaux, sans obligation de résultat et sans qu'aucun garde-fou sur la stratégie de réforme du Gouvernement soit inscrit dans le texte. Il convient donc que le titre du projet de loi reflète cet objectif réel.

Les salariés ont beaucoup perdu ce soir. Le Gouvernement prendra les rênes de l'assurance chômage, à la place des organisations syndicales et patronales, jusqu'au 31 août 2023.

Les allocations chômage seront supprimées après trois refus de CDI. Les abandons de poste seront considérés comme des démissions, sans indemnisation chômage. Les intérimaires qui n'acceptent pas un CDI

qu'il faut forcer à revenir vers l'emploi et qui seraient l'unique cause des maux des entreprises ne trouvant pas de salariés. Nous prenons le problème à l'envers.

Comme la sécurité sociale, l'Unédic est capitale pour les travailleurs, pour notre pays, pour la République ! Il nous faut atteindre le plein emploi pour améliorer le financement de la sécurité sociale et équilibrer le budget de l'Unédic. Aux termes

partenaires sociaux, pour l'évolution de la gouvernance de l'assurance chômage et la négociation des règles d'indemnisation, sur la base d'un document d'orientation. La commission remet donc les partenaires sociaux dans le jeu, contrairement à ce que j'ai entendu dire à plusieurs reprises

abyssal qui existe entre la situation réelle de millions de demandeurs d'emploi et les discours publics, repris ici, qui sont tenus sur eux et, comme toujours, sans eux. Le Gouvernement veut engager une réforme dont le seul résultat sera des milliards

Ensuite, nous avons renforcé le cadre législatif des règles d'indemnisation du chômage en complétant, pour les sécuriser, les dispositifs prévus par le projet de loi, en inscrivant dans le texte le principe de modulation envisagé par le Gouvernement, mais aussi en introduisant des mesures nouvelles, notamment au regard des difficultés de recrutement actuelles.

Enfin, parce que nous sommes encore loin d'avoir atteint le plein emploi, il était particulièrement utile d'améliorer le dispositif de validation des acquis de l'expérience, une initiative portée par le Gouvernement, que nous avons complétée en commission.